À la demande de nos collègues communistes, le Sénat avait débattu en 2014 de l'avenir des colonies de vacances. À cette occasion, j'avais pu insister sur la question de la professionnalisation de l'encadrement, selon moi difficile à imaginer, dans le secteur des séjours collectifs de vacances, divisé entre offre commerciale et fonction sociale, sociétés à but lucratif et organisateurs associatifs, ce secteur n'utilisant près de 150 000 animateurs et directeurs occasionnels que quelques semaines dans l'année, pendant un an ou deux au maximum. J'avais plaidé alors pour que le mode occasionnel, par exemple dans le cadre d'un volontariat de l'animation, puisse demeurer le mode dominant d'encadrement des séjours de vacances, les professionnels n'étant requis que pour la pratique des activités dangereuses ou risquées. Le ministre de l'éducation nationale s'était engagé à poursuivre le dialogue amorcé autour du statut des animateurs et des encadrants et de l'équilibre à trouver entre salariés, volontaires et bénévoles pour offrir à chacun un cadre lui permettant de s'investir dans des projets éducatifs portés par les colonies de vacances, tout en bénéficiant d'un statut protecteur, et de continuer à faire vivre ce creuset d'engagement qu'a toujours été le monde des colonies de vacances. Le constat a été établi et il est partagé par tous, je n'y reviens pas. Nous avons tous en tête également les termes du débat : la question de l'eurocompatibilité, la sécurité des enfants, le code du travail, voire de l'éventuelle fragilisation du champ du volontariat. Néanmoins, nous avons souhaité soutenir la démarche de notre collègue député Hervé Féron et des députés socialistes en reprenant l'amendement portant sur le volontariat d'animation, qui est une forme d'engagement dont ce projet de loi aurait pu traiter, et ce même si cet amendement soulève des difficultés juridiques, nous le comprenons. Le débat à l'Assemblée nationale sur cet amendement a d'ailleurs largement porté sur ces conséquences juridiques.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous indiquer si un groupe de travail a bien été mis en place et quelles sont les avancées sur ce dossier ? Quel est l'avis de la commission ? l'avis de la commission ? Notre collègue évoque un vrai sujet qui concerne non seulement les colonies de vacances, mais aussi les centres de loisirs et les séjours organisés par les communes. Monsieur Magner, vous proposez de créer un volontariat de l'animation

d'examiner une telle réforme, qui a des conséquences juridiques et financières, au détour d'un amendement. Nous n'avons pas d'étude d'impact. Nous n'avons pu, dans le temps qui nous était imparti, mener une analyse approfondie du dispositif ni en discuter avec les acteurs concernés. Tout en reconnaissant la pertinence de votre question, je suis obligée, en l'état de nos connaissances, d'émettre un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

confirment en effet qu'un tel volontariat, même s'il était encadré par le droit national- et nous avons fait toutes les vérifications en l'espèce -serait requalifié en contrat de travail, notamment en raison du lien de subordination qui doit exister entre l'animateur et le directeur de l'accueil. Je ne peux imaginer que soient autorisées des activités d'encadrement d'enfants et d'adolescents ne s'inscrivant pas dans un régime de responsabilité hiérarchique à même de garantir la sécurité. Aucun parent n'accepterait que son enfant soit confié à des personnes qui ne respecteraient pas un lien hiérarchique avec le directeur du centre. Certes, l'histoire des accueils collectifs de mineurs s'inscrit dans une logique d'animation volontaire. Mais je vous rappelle que, dans le vaste secteur des loisirs éducatifs, coexistent, parfois au sein d'une seule et même structure, des approches et des pratiques qui ne sont pas toujours exemptes d'une logique commerciale. J'attire donc votre attention sur le fait qu'un tel statut, s'il était créé, serait requalifié et constituerait une brèche irréformable. Celle-ci aurait des incidences directes sur les différentes formes de volontariat que nous connaissons aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'engagement de service civique- nous ne voulons pas que le service civique puisse être ouvert aux centres d'accueil de mineurs - , des volontariats internationaux ou du service volontaire européen. Mon souhait, monsieur le sénateur, est de ne pas créer de confusion entre le volontariat et le salariat, de ne pas fragiliser l'ensemble de l'édifice que nous avons construit en matière de volontariat. J'ai procédé à des consultations et nous estimons que la solution ne passe pas par le volontariat de l'animation. Il faut trouver Il faut trouver une autre formule pour valoriser ces centres d'accueil et ces colonies de vacances. C'est la raison pour laquelle je sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.

sur l'article. Soyons clairs : aujourd'hui, le dispositif est vu comme un palliatif au chômage, manquant son objectif fondamental d'engagement civique. Tout ce qui aurait pu le sécuriser et le distinguer d'un emploi a été, selon moi, rejeté au nom même de cette non-substitution. Ainsi, être en service civique aujourd'hui, c'est parfois effectuer quarante-huit indemnisées 573 euros, dont 106 euros à la charge de la structure, sans cotiser pour les droits sociaux et sans bénéficier des acquis des salariés. Et ce n'est pas le manque budgétaire continu de l'Agence du service civique qui permet de lutter contre ce phénomène, comme l'a rappelé son président, Yannick Blanc, il y a quelques semaines en audition.

au centre de consultation », ou « maîtrise d'une langue étrangère exigée », ou « nous recherchons un profil expérimenté ou diplômé du supérieur » ... Les annonces de cet acabit m'ont beaucoup étonnée. Je considère- et on en avait déjà parlé l'année dernière -que l'objectif du service civique, c'est partir partir du projet du jeune et aider celui-ci à aller plus loin dans son projet. On en vient donc à se demander quel est l'objectif d'une généralisation du dispositif et dans quelle mesure cela devrait permettre d'éviter les abus et d'améliorer qualitativement les missions.

En effet, il faut se prémunir contre le risque d'un grignotage du secteur des stages et des premières expériences professionnelles. Quelques dérives seraient à craindre à ce sujet. Avec le service civique, les jeunes sont accompagnés dans le cadre d'un projet qui leur permet de valoriser leurs compétences et leur expérience, ainsi que de structurer leurs savoir-être et Le service civique ne doit pas remplacer un emploi, il doit préparer un jeune à être embauché. Cette indication manque à ce texte pour se limiter à l'aspect social de l'encadrement et à l'intégration par la découverte. L'ensemble de ce texte est construit pour veiller à l'égalité des chances des différentes catégories à la recherche d'un emploi. Étant donné que le service civique concerne des jeunes de 16 à 25 ans qui n'étudient plus, nous approuvons le fait que ne soit pas exigé le

En ce sens, ouvrir, par cet article, la possibilité pour des entreprises publiques ou des offices d'HLM d'accueillir des volontaires en service civique, c'est courir le risque, évidemment, de dénaturer la dimension citoyenne et civique de ce dispositif. Cette mesure peut s'avérer contraire à la volonté affichée par le Gouvernement de valoriser l'engagement citoyen et de rendre imperméable la frontière entre emploi, d'un côté, et service civique, de l'autre. Le second problème, c'est que, au final, cette mesure peut constituer aussi un frein à l'emploi, en encourageant des entreprises à recourir, de manière quelque peu abusive, à des volontaires en service civique, rémunérés à hauteur de 106 euros par l'entreprise. Sans ouverture de protection sociale et avec une très faible rémunération, le service civique ne peut constituer, en tout cas à nos yeux, un outil de mise en concurrence entre jeunes en recherche d'expérience et salariés en emploi ou en recherche d'emploi. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article

de la structure qui l'accueille. Notre commission a étendu la liste des organismes susceptibles d'accueillir des volontaires en service civique de faire face à l'objectif du Gouvernement d'accueillir la moitié d'une classe d'âge en service civique, soit 350 000 jeunes,

Quel est l'avis du Gouvernement ?

L'objectif ambitieux que nous nous sommes fixé sera atteint en tenant compte d'une exigence : ne pas altérer la qualité des missions qui sont proposées, tout en étendant le nombre de structures qui pourront accueillir des volontaires. Un exemple : le palais de Tokyo souhaite développer un programme de service civique, mais ne peut être agréé, car il est constitué sous la forme d'une société détenue à 100 % par l'État. l'article 10 devait être supprimé, cela rendrait impossible l'agrément qui est proposé dans le texte que j'ai l'honneur de défendre devant la Haute Assemblée. Le fait que ce critère d'éligibilité soit rempli ne préjuge pas pour autant que les missions proposées par ces organismes seront agréées par l'Agence du service civique.

qui sont aujourd'hui en flux, il n'y a pas, ici ou là, de possibles abus, mais nous sommes là pour les corriger. En tout cas, la volonté politique est réelle en la matière. Compte tenu de l'ensemble de ces verrous, monsieur Favier, je considère que votre amendement ne peut être retenu. J'émets

à M. Maurice Antiste. Le service civique a pour but de soutenir l'engagement dans la vie citoyenne et de renforcer la place des jeunes dans la République. Si favoriser l'engagement dans les associations et les organismes sans but lucratif répond clairement à cet objectif, la mise à disposition d'engagés du service civique au sein des organismes d'habitation à loyer modéré, de sociétés publiques locales ou de sociétés dont l'État détient la totalité du capital ne semble pas atteindre ce but. En outre, étant donné les missions accomplies par ces organismes et ces sociétés, la mise à disposition d'engagés du service civique permettrait à l'organisme et auxdites sociétés de bénéficier d'une main-d'oeuvre à bas coût.

En effet, l'article 10 vise à élargir le champ des structures pouvant recourir au service civique, notamment en y intégrant les organismes de logement social, les OLS, qui regroupent à la fois les offices, les SA HLM et les

s'agit nullement des SEM dans leur globalité. Dans la mesure où les SEM ont pleine capacité juridique et que leurs statuts sont les mêmes

totalement par le privé. Ce sont en général des entreprises de travaux publics qui sont actionnaires de ces SA HLM, alors que les SEM ont en majorité

Le service civique a en effet pour objectif de permettre à des jeunes souhaitant s'engager dans des missions d'intérêt général de pouvoir intégrer des structures qui proposent ce type d'actions.

structures déjà proposées dans le projet de loi. Ces sociétés, comme leur nom l'indique, sont des structures de l'économie sociale et solidaire qui associent des acteurs sur un territoire, avec comme objectif de produire des biens ou des services qui présentent un intérêt collectif.

Le service civique, je le rappelle, est un engagement volontaire d'un jeune pour accomplir des missions à valeur sociale, voire républicaine. Il ne faut en aucun cas confondre cette mission avec un emploi. emploi. Nous n'avons pas pris en considération simplement le statut des structures pour considérer qu'elles pouvaient accueillir des volontaires en service civique, mais nous nous sommes intéressés de près aux missions qu'elles pouvaient proposer, et c'est pourquoi nous avons élargi

des sociétés publiques locales ne conduisent à des abus. En revanche, nous avons rejeté la possibilité pour des organisations internationales dont le siège est implanté en France d'accueillir des volontaires en service civique, estimant que le risque de substitution

n'y avait pas de place pour des missions à caractère social ou républicain en leur sein. Nous les avons donc écartées pour éviter tout risque de substitution à un emploi.

clair et précis, ces sociétés ne sont pas comprises dans le champ de l'article 10 du projet de loi, qui ne vise que les organismes d'habitations à loyer modéré. Ces amendements permettent de les inclure dans le champ des organismes qui peuvent recevoir un agrément,

service civique à des organismes qui ont un caractère commercial, même s'il s'agit de sociétés coopératives. Il est préférable de viser, comme le texte le fait déjà, les entreprises

Il est plus que jamais nécessaire, nous le savons, de recréer un creuset social, afin que l'idée de la République et ses valeurs vivent pour tous les citoyens. Le service civique doit être ce lieu de rencontre avec la République concrète et vivante. l'article 10 étend aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux sociétés publiques locales et aux sociétés dont l'État détient la totalité du capital la possibilité d'accueillir des volontaires en service civique. Le présent amendement vise à étendre encore le nombre de structures agréées pour le service civique. Il a pour objet de permettre que des structures politiques accueillent des jeunes en service civique. Dans ces structures, le risque de substitution des missions des volontaires à un stage ou un emploi paraît moins important. Pourtant, les partis, notamment, sont un outil essentiel de la démocratie de la vie civique. Alors que la vie politique souffre d'un fort discrédit parmi les jeunes, qui sont fortement touchés par l'abstentionnisme, l'accomplissement d'un service civique au sein d'une structure partisane pourrait permettre de recréer du lien entre la jeunesse et les partis politiques. Le jeune qui ferait son service civique au sein d'un parti découvrirait la vie militante, la vie politique et le fonctionnement des institutions. Et, nous le savons, cette expérience peut être un tremplin important, du fait de la diversité des fonctions exercées et des sujets traités. De nombreux étudiants dans les instituts d'études politiques, les IEP, effectuent de tels stages. La citoyenneté est avant tout une pratique, qu'il s'agit de faire vivre ou revivre. Tel est l'objet de cet amendement.

effet, s'engager pour la Nation, c'est une manière aussi de s'engager en politique au sens le plus large du terme. Mais le service civique ne doit pas être le remède au désengagement politique des jeunes, notamment à l'abstention, malheureusement trop importante. Je terminerai mon propos par un argument plus juridique

cette mesure semble être une réponse adaptée à un problème réel, celui de l'utilisation des services civiques par certaines structures peu scrupuleuses. Offres de missions correspondant à des emplois déguisés, recours systématique et massif à des volontaires sous-encadrés : les cas sont assez nombreux dans lesquels une inscription en amont sur le registre unique du personnel aurait permis d'alerter l'Agence du service civique, monsieur le ministre. Cette mesure doit être appréhendée non pas comme une sanction, mais comme une volonté de transparence. Les conditions d'un service civique réussi tiennent autant d'une mission d'intérêt général enrichissante que d'un encadrement suffisant par des tuteurs formés. Malheureusement, le service civique est parfois encore considéré comme une solution pour endiguer un sous-effectif chronique ou éviter le recours à une embauche autrement plus coûteuse, le tout au mépris de l'esprit du dispositif, des conditions d'accueil des volontaires, mais aussi des conditions de travail des salariés.

La commission spéciale a supprimé l'article 11 , qui prévoyait l'information des représentants du personnel sur les volontaires en service civique, au double motif qu'introduire des dispositions relatives au service civique dans le code du travail serait source de confusion et que le contrôle du service civique relèverait de l'État, et non des partenaires sociaux. Nous ne partageons pas le premier point de cette analyse : garantir la non-substitution du service civique à l'emploi n'implique pas que les acteurs du champ professionnel doivent en être tenus à l'écart que les dispositions relatives au service civique soient tenues éloignées du code du travail. Sur le second point, certes, le contrôle incombe à l'Agence nationale du service civique, et non aux partenaires sociaux, mais ceux-ci peuvent jouer un rôle d'alerte pour une meilleure efficacité de l'Agence. C'est pourquoi nous souhaitons rétablir l'information des représentants syndicaux dans les entreprises et administrations. En outre, la montée en charge du service civique ne va pas se faire dans les petites associations bénéficiaires du chèque emploi service, non tenues au registre unique du personnel, mais dans les nouvelles structures ouvertes à l'agrément et le secteur public. C'est pourquoi nous proposons le rétablissement de l'article 11 .

Considérer les syndicats comme des lanceurs d'alerte à l'égard de structures habilitées à accueillir des jeunes en service civique qui seraient

Introduire un lien avec le code du travail, alors que l'on a bien dit qu'il n'y avait pas de lien de subordination, me semble contraire à l'esprit du dispositif, dès lors que l'on a pris toutes les précautions.

ont recours au chèque associatif et, dans ce cas, elles sont dispensées de tenir ce registre unique du personnel. Dès lors, comment vont-elles faire et comment allez-vous gérer cette situation,

Globalement, une structure agréée pourrait « prêter » des volontaires sous sa responsabilité à une structure non agréée, mais qui pourrait l'être si elle le demandait. Plusieurs questions Pourquoi la structure non agréée, dans la mesure où elle veut accueillir des volontaires, ne fait-elle pas sa demande d'agrément ? Cela serait autrement plus simple et transparent.

Par ailleurs, j'admets être surprise. À l'Assemblée nationale, le rapporteur du texte, M. Hammadi, explique que l'intermédiation est amenée à disparaître et, pourtant, on l'inscrit dans la loi

Mais en parallèle, il prend le risque, par l'intermédiation, que certaines structures d'accueil ne deviennent de véritables boîtes d'intérim de volontaires, qui seraient des plates-formes de transition pour des personnes précaires en mission de service civique, mais occupant en réalité des emplois déguisés. Je vous remercie,

les modalités par lesquelles un volontaire pourrait être mis à la disposition de personnes morales de droit étranger, afin de développer les missions de service civique à l'international. Nous souhaitons ainsi mettre en oeuvre une forme de droit à la mobilité internationale. Aujourd'hui, le dispositif d'intermédiation ne permet pas de mettre à disposition des volontaires auprès de structures étrangères, alors même

que peuvent revêtir ces structures étrangères, l'amendement du Gouvernement prévoit de viser spécifiquement les collectivités territoriales étrangères et les organismes sans but lucratif de droit étranger, ce qui permet de sécuriser le dispositif et d'éviter toute dérive,

commission met en garde contre le fait que de nombreux jeunes volontaires se verraient confier des missions qui s'apparenteraient davantage à une forme d'emploi déguisé, venant pallier les manques d'effectifs de la structure d'accueil, qu'à une véritable mission d'intérêt général au service de la collectivité. Des défaillances dans la qualité de l'accompagnement de la mission sont également envisageables. C'est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet de prévoir un renforcement des obligations de la structure intermédiaire. Il s'agit de s'assurer qu'elle a les capacités de remplir, de manière satisfaisante, les missions que l'Agence du service civique lui délègue de fait.

Monsieur le ministre,

spéciale. Il a pour objet d'organiser les modalités par lesquelles le représentant de l'État dans le département anime le développement du service civique à l'échelon local, dans le respect absolu du principe de libre administration des collectivités territoriales. D'ailleurs, il m'a semblé qu'un candidat à la primaire de la droite et du centre pourrait remettre en cause ce principe, ce que je regretterais naturellement

reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel doivent être présentes au nombre de ces acteurs. Le respect du principe de non-substitution à l'emploi, évoqué à plusieurs reprises dans cet hémicycle et réaffirmé avec force dans le projet de loi, implique d'associer

concerne l'amendement n° 244, vous l'aurez compris, le Gouvernement est favorable à la réintroduction des organisations syndicales dans la gouvernance locale. Toutefois, la rédaction de l'amendement du Gouvernement, qui clarifie le rôle de chaque partie, nous semble plus appropriée. Le même amendement prévoit, en outre, de définir une durée hebdomadaire moyenne d'activité de 24 heures par semaine. Les associations partenaires de la mise en oeuvre du service civique, qui proposent aujourd'hui plus de 70 % des missions, sont divisées sur une modification de ce paramètre. Les modalités doivent rester souples et, là aussi, efficaces, pour que le dispositif puisse s'adapter aux différentes formes de missions qui sont proposées aux jeunes. Nous sommes dans une phase de montée en charge du service civique et je ne suis pas favorable

Au fur et à mesure de l'histoire, cela change. Au XIX siècle, beaucoup de travailleurs sociaux étaient bénévoles.

Ce serait une erreur de ne pas parler de ce sujet avec les organisations syndicales, qui peuvent très bien comprendre que certaines tâches relèvent du service civique, cependant que d'autres relèvent du salariat. Vouloir éviter d'en parler me paraît une puissante erreur

Cet amendement vise à créer de nouvelles protections pour les volontaires en service civique. Cela doit, à nos yeux, s'articuler autour de deux axes fondamentaux : étanchéifier la frontière entre l'emploi et la mission de service civique, tout en impliquant les salariés dans le processus. Ces deux ambitions peuvent paraître contradictoires, certes, mais sont en fait complémentaires pour deux raisons très simples. Première raison, le volontaire du service civique, présent dans les structures et encadré par des salariés, côtoie de fait le monde du travail dans le cadre de sa mission. Seconde

En réintégrant les syndicats de salariés dans la gouvernance territoriale du service civique tout d'abord. Il s'agit de faire notamment entendre la voix des tuteurs dans la coordination du dispositif. Le second aspect, c'est de limiter le nombre de volontaires par structure, afin d'éviter les situations dans plus de volontaires que de salariés-tuteurs, ce qui nuit à la bonne exécution de la mission. Notre dispositif, calé sur celui qui concerne les stages et qui est prévu dans le décret du 26 octobre 2015, doit permettre d'éviter que le recours aux volontaires ne soit le réflexe pour pallier un besoin chronique

à 35 heures, voire 48 heures sur une durée maximale de six jours en cas de dérogation. Ces dérogations, accordées en cas d'excès d'activité sur une période donnée, ne donnent droit à aucun congé après la période de suractivité

engagement bénévole. Il s'agit aussi et surtout de renforcer la distinction entre service civique et emploi. Cela ne peut se faire que si la durée du service civique ne dépasse pas, en moyenne, 24 heures

à rappeler qu'en aucun cas le service civique n'est un emploi : il s'agit d'un engagement dans la vie d'un jeune, au même titre qu'un engagement dans une association. association. Compte tenu de cette absence de consensus sur la validation d'une règle plutôt qu'une autre, je propose d'en rester à la règle actuelle, qui impose un minimum de 24 heures. Il faut un minimum, parce que le jeune doit vraiment s'engager et découvrir la réalité des choses. Enfin, je félicite le groupe CRC de son extrême précision dans la définition d'un quota d'accueil de jeunes en service civique. Mes chers collègues, j'ai bien compris votre souhait de préserver un accueil de qualité, mais il ne me semble pas opportun

et en volontariat international à la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours de troisième voie. Or les rédactions actuelles

Or les rédactions actuelles des articles 12, qui touche au code du service national, et 36, dont je parlais à l'instant, et qui touche aux lois portant dispositions statutaires dans la fonction publique, ont pour conséquence d'exclure ces deux sortes d'engagement des expériences exigées pour se présenter à ce type de concours de la fonction publique. Il n'est pas logique, mes chers collègues, que ce qui est possible pour les concours internes ne le soit pas pour les concours de troisième voie, qui, je le rappelle, reposent sur l'expérience acquise, d'autant qu'une expérience au service de l'intérêt général est

Le présent projet de loi reprend ce principe et le conforte. Il s'agit d'ailleurs, me semble-t-il, d'une disposition déjà très avantageuse pour les personnes concernées. À titre d'exemple, les années passées en apprentissage auprès d'une personne publique permettent seulement l'inscription au troisième concours, qui propose, en règle générale, moins de places que le concours interne. L'amendement prévoit que le service civique et le volontariat international permettent également de s'inscrire au troisième concours. Je n'y suis pas du tout favorable, car cela autoriserait une « double inscription » aux concours internes et aux troisièmes concours, créant ainsi une inégalité par rapport à l'apprentissage, seulement éligible au troisième concours, comme je viens de le souligner. Enfin, je rappelle que le troisième concours s'adresse aux personnes ayant une activité professionnelle dans le secteur privé et que le service civique est un engagement citoyen, pas une activité professionnelle au sens strict du terme.

Quel est l'avis du Gouvernement ? L'article 36 du projet de loi, qui comprend plusieurs mesures relatives à la fonction publique et que nous retrouverons lors de l'examen du titre III, et notamment sur le troisième concours, prévoit la prise en compte du service civique dans la période nécessaire pour s'y présenter.

Si la reconnaissance législative des cadets de la défense peut s'entendre, la réforme qui est proposée me pose deux problèmes. Tout d'abord, alors que le dispositif implique aujourd'hui directement l'éducation nationale dans le cadre de parcours scolarisés, plus rien n'est prévu à cet égard, et l'on confie à l'armée la mission d'un enseignement moral et civique. Je m'étonne de retrouver ici une mesure reprise d'une proposition de loi de Marianne Dubois et Laurent Wauquiez tendant à retirer ses prérogatives à l'éducation nationale pour les donner à l'armée.

Second problème de taille : l'avancement de l'âge auquel les enfants participeraient au dispositif. Alors que sont concernés aujourd'hui des adolescents d'au minimum quinze ans, le texte prévoit de l'ouvrir aux enfants dès douze ans,

d'aller à la rencontre de militaires et d'unités combattantes. Ces enfants, qui choisissent librement ce parcours, en sont plutôt très satisfaits. Vous proposez d'associer le ministère de l'éducation nationale à la mise en oeuvre du programme des cadets de la défense et de porter l'âge minimal des jeunes participants de douze à seize ans. Avec tout le respect que je dois au ministère de l'éducation nationale,

Ensuite, s'agissant d'un programme de jeunesse offrant aux jeunes de pratiquer diverses activités culturelles et sportives- cela ressemble plus au scoutisme qu'à une activité militaire -et de recevoir un enseignement moral et civique complémentaire, il serait contre-productif de le limiter aux jeunes de seize ans et plus, alors que ce projet de loi a pour ambition d'encourager et de développer l'engagement civique chez les plus jeunes.

Le principal obstacle auquel se heurte aujourd'hui le programme des cadets est l'absence totale de pilotage national et de crédits budgétaires dédiés ». Le projet de loi répond à la question du pilotage, puisqu'il est précisé que le programme est mis en oeuvre par le ministère de la défense. En revanche, demeure le problème de financement.

Il s'agissait alors de financer les tenues des cadets et le transport de leurs collèges respectifs jusqu'à la base aérienne, ce qui représentait une somme d'environ 5 000 euros pour une année de fonctionnement et une quinzaine de cadets. C'est loin d'être une somme astronomique et, pourtant, sans l'aide parlementaire, l'opération n'aurait pas vu le jour, car la base aérienne, qui mettait à disposition ses locaux et ses réservistes, et l'éducation nationale, qui impliquait les principaux des collèges pour l'organisation et le choix des cadets, n'avaient aucun budget en propre pour la mener. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles seront les orientations budgétaires pour l'année prochaine afin de faire vivre ce dispositif ? Concernant l'amendement porté par nos collègues du groupe CRC, nous ne pensons pas qu'il faille changer à ce stade les modalités du dispositif des cadets de la défense. Voilà

Créé par la loi du 10 mars 2010 dans un large consensus politique, le service civique peut connaître aujourd'hui une nouvelle étape.

Je reconnais qu'en déposant mes deux propositions de loi, en 2006 et en 2015, je visais à mettre en place un service civique obligatoire, composé de deux périodes étalées dans le temps.

pour une durée maximale de trois ans. Mes chers collègues, plutôt que de refuser le service civique universel, mettons en place une expérimentation, et nous pourrons ensuite juger si ce dispositif est une bonne chose ou s'il s'agit d'une mauvaise idée. Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Les obstacles sont-ils insurmontables ? Quel pourrait en être le coût ?

mérite de survivre à cette soirée pour être éventuellement reprise dans les prochains mois, puisque des débats politiques extrêmement importants

votre proposition, à suivre l'actualité électorale des prochains mois et à continuer à pousser votre idée. En attendant, j'émets un avis défavorable.

désiré par les jeunes. À mon sens, cet objectif de 800 000 missions de service civique est aujourd'hui inabordable pour notre pays. Je vous demande de l'intégrer non pas comme une contrainte, mais comme une réalité objective. Par définition,

conscrits potentiels passant au travers des mailles du filet. Je n'ai pas envie d'avoir un service civique universel et obligatoire qui aboutirait à ce type de résultat, ce qui ne serait bon pour personne. Le Président

L'idée d'un service civique obligatoire universel pourrait aussi conduire à raccourcir la durée du service civique à quelques mois, ce qui serait totalement contradictoire avec l'objectif initial de la loi de 2010. Vous l'aurez compris, monsieur le sénateur, je suis au regret que je ne vois pas l'intérêt d'une expérimentation en la matière. J'émets donc un avis défavorable, ce qui n'est pas pour vous une surprise.

on privilégie malheureusement un peu trop souvent l'aspect financier, alors que tout relève de l'humain, je me rallierai naturellement à l'avis des rapporteurs de la commission, qui ont beaucoup travaillé sur

courtoisie de considérer que l'avis émis par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale devait être respecté.

J'attire votre attention sur le fait que le groupe Les Républicains, qui est, comme vous le savez, le plus important de notre assemblée, a été frappé 15 fois par les rigueurs de l'article 45,

Le projet de loi tend à valoriser l'engagement des étudiants. Or il conviendrait, pour donner corps au parcours citoyen, de ne pas attendre les études supérieures, lesquelles ne concernent pas toute une classe d'âge, pour valoriser l'engagement. Qu'il s'agisse du bénévolat associatif, de la participation à la réserve opérationnelle, du volontariat en tant que sapeur-pompier ou du service civique, toutes ces formes d'engagement sont accessibles dès 16 ans ; elles doivent donc être reconnues et valorisés plus tôt. Quant au volontariat dans les armées, s'il s'adresse à des majeurs, il doit pouvoir être valorisé en cas de reprise d'études secondaires, le service militaire volontaire concernant prioritairement les jeunes peu ou pas diplômés.

Nous avons mis en place l'enseignement moral et civique ; nous développons le parcours citoyen généralisé, matérialisé par le livret citoyen. Nous bénéficions de bénévoles prêts à agir dans nos établissements, dans le cadre de la réserve de l'éducation nationale. Quelle articulation, quelle synergie, entre ces dispositifs, pour une citoyenneté en actes dès le plus jeune âge ? Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la teneur du livret citoyen, qu'il est question de délivrer à partir de 16 ans. Pourquoi attendre la fin de la scolarité obligatoire, d'autant que le parcours citoyen débute, quant à lui, dès l'école primaire ?

Je rappelle que, au-delà du baccalauréat, nous avons voulu mettre en valeur l'engagement spécifique des jeunes tout au long de leur parcours. Tel est le cas avec le parcours citoyen dans le système scolaire, qui se prolongera demain avec la mise en place du livret citoyen, annoncé par le Président de la République. Lorsque cet engagement est substantiel, reconnu

L'engagement serait-il réservé aux étudiants en BTS, en licence, en master ou en école d'ingénieurs ? Peut-être un docteur n'a-t-il pas intérêt à valoriser les aptitudes qu'il aurait développées dans un engagement citoyen ? Celles-ci seraient-elles inutiles pour mener une carrière d'enseignant ou de chercheur ? Dans la recherche d'un emploi, les docteurs sont confrontés à la concurrence, comme les autres diplômés de l'enseignement supérieur. L'enquête du CEREQ sur la génération de diplômés de 2007 montre que le taux de chômage des docteurs reste plus important que celui des ingénieurs trois ans après l'obtention de leur diplôme, que 40 % d'entre eux travaillent dans le secteur privé et 32 % en dehors du domaine de la recherche.

serait une insulte au plus haut diplôme de notre pays, et entraînerait la délivrance de doctorats à des personnes qui n'auraient pas fait de recherche, donc de doctorats au rabais.

La reconnaissance des compétences acquises hors cursus ne sera qu'un complément. Depuis plusieurs années, nous travaillons à la valorisation du diplôme de docteur, formation professionnelle à la recherche, formation professionnelle par la recherche. L'ouverture d'esprit et la pratique de ses détenteurs sont vantées pour leur permettre d'accéder à d'autres emplois que ceux de la recherche ou de l'enseignement, qui ne peuvent recruter tous les diplômés, dont le nombre croît chaque année.

monsieur le ministre, Le Gouvernement s'était opposé à une telle exclusion lors des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale. En effet, les dispositions de l'article 14 permettent aux étudiants de valider, au titre de leur formation, les compétences qu'ils acquièrent dans le cadre d'activités extra-académiques. Madame la rapporteur, il ne s'agit pas de délivrer le diplôme du doctorat à un étudiant « engagé ». Mais il peut s'agir de le dispenser, par exemple, de tout ou partie des formations complémentaires proposées par l'école doctorale dans le cadre de son cursus et de les faire valoir dans le portfolio de compétences valorisant l'ensemble des acquis en fin de doctorat.

La constitution d'un portfolio de compétences est utile, et le sera de plus en plus pour asseoir un parcours professionnel et crédibiliser les aptitudes recherchées pour telle ou telle mission. exclure le diplôme de doctorat de cette démarche est une erreur profonde, qui ne peut que desservir les doctorants, qui ont eux aussi besoin de se frotter à la vie réelle et d'en faire la démonstration au travers du portfolio de compétences évoqué par M. le ministre.

apport de nouvelles compétences, capacité d'adaptation, ouverture d'esprit -, celui pour l'entreprise est moins souvent perçu, il faut le reconnaître. Or les connaissances et compétences acquises par un jeune pendant la période de mobilité constituent également des atouts indéniables pour la compétitivité des entreprises. Cela participe également de leur image de marque, et certaines s'en réclament d'ailleurs, et ce à juste titre. Tous les jeunes qui partent à l'étranger ne sont pas des jeunes qui ne reviennent pas travailler en France ! La suspension du contrat de travail prévue pendant la période de mobilité déséquilibre les conditions d'une mobilité réussie et crée une insécurité juridique pour les apprentis. Je pense notamment à l'absence de couverture sociale professionnelle, à l'impossibilité de se prévaloir de l'expérience acquise dans le cadre de la certification,

et de formation. Aussi, il est proposé de substituer aux dispositions de l'article 14 A des dispositions nouvelles, qui sont de nature à soutenir véritablement le développement de la mobilité internationale, notamment en élargissant les possibilités de mobilité au-delà de l'Union européenne, ou encore en ouvrant la possibilité aux OPCA,

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 46 amendements au cours de la journée